Monsieur le président,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

En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable- 16 voix pour, aucune voix contre -à la nomination de M. Antoine Petit à la présidence du Centre national de la recherche scientifique.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 L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, créée sur l'initiative du groupe Les Républicains, en application du droit de tirage prévu par l'article 6 du règlement.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 L'ordre du jour appelle la désignation des membres du groupe de travail préfigurant la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance.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 Il appartiendra au Sénat de transformer ce groupe de travail en commission spéciale, après la transmission du projet de loi, conformément à l'article 16 de notre règlement.

que les interventions publiques des membres du G20. Pourquoi des crises ? Leur moteur, c'est l'abondance de liquidités, de monnaie, qui stimule bulles financières et prolifération de créances douteuses. Lorsque ces bulles crèvent, les circuits financiers coagulent. Et quand domine, comme aujourd'hui, un oligopole de banques géantes à vocation mondiale interconnectées à la vitesse de la lumière, c'est le fonctionnement du système tout entier, et de l'économie avec lui, qui est bloqué. À l'origine de la liquidité, on trouve la création monétaire des banques, centrales et, surtout, commerciales. Dans les économies financiarisées comme la nôtre, le crédit et l'endettement deviennent le carburant du système et la spéculation l'activité principale des établissements financiers. Dix ans après la grande crise de 2007-2008, après treize G20, l'intervention financière massive des États et des banques centrales, un entassement de projets de réformes, force est de constater que le système financier est toujours aussi dangereux. loin de diminuer, le volume des liquidités en circulation a explosé. Stimulé par une politique de taux bas, voire négatifs, l'endettement public et privé n'a cessé d'augmenter. Alimenté par les politiques de des banques centrales, le stock de liquidités a fait de même. Ainsi, en zone euro, si l'endettement public est repassé sous la barre des 90 % du PIB- 96 % pour la France -, l'endettement privé en représente 170

D'où la formation de bulles spéculatives sur les obligations, les actions des entreprises américaines, sur l'immobilier dans la plupart des grandes villes. Deuxièmement, l'oligopole bancaire- plus de 50 000 milliards de dollars d'actifs en 2012, soit 70 % du PIB mondial -est toujours « trop gros pour faire faillite ». La France y tient son rang : le bilan de BNP Paribas- 2 077 milliards d'euros en 2016 -tangente le PIB national. Avec ceux de la Société générale, du Crédit agricole et de BPCE, on atteint trois fois le PIB français. En Europe, les graves difficultés d'établissement systémiques, comme HSBC, Crédit Suisse et, surtout, Deutsche Bank, la plus grande banque d'Allemagne, inquiètent. Quant aux banques européennes plus modestes, le total des créances douteuses plombant leurs bilans se situerait entre 1 000 milliards et 1 200 milliards d'euros, dont 300 milliards pour l'Italie. Troisièmement, la régulation est toujours « ni faite ni à faire ». Faute de temps, je me limiterai à la question de la séparation entre banques de dépôt et banques d'affaires et à la question des ratios de fonds propres exigibles. Les idées qui ont été mises sur la table par Michel Barnier sont des idées [ ...] irresponsables et contraires aux intérêts de l'Union européenne » : cette charge de Christian Noyer, alors gouverneur de la Banque de France contre le commissaire européen français est révélatrice de l'enthousiasme des banquiers européens pour la séparation bancaire

Conclusion de ce trop rapide survol de dix années de crise financière et de stagnation économique : la probabilité de réédition d'un nouveau krach n'a pas diminué. Tous les ingrédients- certains sous une forme nouvelle -sont toujours là.

au point que la BCE a relevé son taux directeur. Vous connaissez la suite. À ce jour, le monde de la finance retient son souffle, attendant l'arrêt de la perfusion de liquidités des banques centrales et la remontée des taux. Ce qui adviendra, on le sait d'autant moins que, selon la formule d'Henri Sterdyniak, nous connaissons, depuis 2010, « une instabilité stable qui n'a aucune rationalité. Elle est insoutenable et, paradoxalement, le système tient bon ». Le système financier peut-être, mais pas forcément les nerfs de ceux qui, pâtissant toujours de ses dégâts et de l'attentisme politique général, ont transformé les élections en « émeutes électorales » : forte poussée de l'extrême droite partout en Europe, séparatismes nord-italien et catalan, Brexit, élection de Donald Trump aux États-Unis, explosion de l'abstention en France. élection présidentielle, le candidat élu contre celui de l'extrême droite n'a rassemblé que 43,6 % des inscrits, l'abstention et les votes blancs ou nuls, 34 %.

Du jamais vu pour une consultation de cette importance ! Comment ne pas voir dans cette dissidence et ces « émeutes électorales » un désaveu du système tel qu'il fonctionne ? Or, comme l'histoire l'a montré, un système démocratique ne saurait survivre à la perte de sa légitimité. Les financiers, dans leur patois, appellent cela le « risque politique ». Mais qui a bien pu dire que gouverner, c'était prévoir ?

Analyser le passé est toujours utile ; c'est l'occasion de nous interroger sur notre action, mais aussi de l'éclairer, en répondant aux questions qu'elle peut soulever. En ce sens, même si nous ne partageons pas toujours les conclusions de votre rapport, monsieur le sénateur, le travail important que vous avez réalisé est très apprécié. Votre rapport évoque beaucoup de sujets, mais je souhaiterais revenir sur trois points qui me semblent mériter un éclairage particulier particulier : les actions mises en place pour renforcer le système bancaire ; la nécessité de renforcer la zone euro pour éviter qu'une crise comme celle des dettes souveraines ne se reproduise enfin, les questions d'inégalité, qui sont au coeur de votre rapport et de vos préoccupations. Vous vous interrogez, dans ce rapport, sur la solidité de notre système bancaire. C'est une question essentielle, qui a toute notre attention. Depuis la crise, nous avons oeuvré, en lien avec nos partenaires étrangers, pour que les banques aient les ressources nécessaires pour absorber les pertes éventuelles, pour être en capacité de se recapitaliser sans exposer les finances publiques et pour faire face à des aléas de marché. Ainsi, concernant le renforcement de la solvabilité des banques, les exigences de Bâle ont, par exemple, doublé les niveaux de fonds propres minimum requis depuis 2011. Les six plus grandes banques françaises ont désormais un ratio de solvabilité agrégé de 13,2 % fin 2016, contre 5,8 % en 2008. Ce mouvement de renforcement des fonds propres, et donc d'accroissement de la résilience, se retrouve dans les autres systèmes bancaires européens et mondiaux. Il se double d'un renforcement de la qualité de ces fonds propres, ainsi que d'un accroissement des exigences afin de tenir compte de l'ensemble des risques identifiés au bilan, mais aussi des risques potentiels. Au niveau européen, la mise en place de l'union bancaire constitue une étape essentielle permettant une meilleure supervision des banques. L'ensemble du secteur bancaire a par ailleurs fait l'objet d'un examen de la qualité des bilans et a été soumis à des tests de résistance. Enfin, l'Union européenne s'est dotée d'un instrument très ambitieux de résolution des crises bancaires, dont la philosophie est de disposer d'outils permettant de garantir qu'en cas de pertes celles-ci seront portées par les actionnaires, voire les créanciers, tout en protégeant les déposants et les finances publiques. un rôle moteur dans l'achèvement de l'Union bancaire, qui appelle encore des décisions faisant l'objet de discussions en cours. Vous vous interrogez également sur la capacité de la zone euro à résister aux crises et sur sa pérennité. Je tiens à rappeler que l'euro est un projet économique et politique inédit, qui a doté l'Europe d'une monnaie stable et crédible. Cette monnaie est utilisée quotidiennement par près de 340 millions de personnes dans 19 États membres. C'est la deuxième devise la plus importante dans le monde, avec le quart des réserves de change. La crise de la zone euro a toutefois mis en évidence des lacunes dans son fonctionnement, qui ont été pour partie comblées. Ainsi, d'importantes évolutions ont déjà été réalisées, notamment pour promouvoir la stabilité financière au sein de la zone- je pense notamment à la création de mécanismes de gestion de crises des dettes souveraines et bancaires. Le Président de la République et le Gouvernement restent convaincus que le renforcement de la zone euro est la meilleure façon de prévenir les crises futures. Parmi nos priorités pour avancer dans ce domaine, nous défendons une plus forte intégration financière par l'achèvement de l'Union bancaire et la mise en place d'une véritable union des marchés de capitaux. l'amélioration de nos instruments de gestion de crise, en renforçant le mécanisme européen de stabilité, ainsi qu'une plus forte intégration économique et, à plus long terme, la mise en place d'une capacité budgétaire propre à la zone euro permettant aux États de mieux faire face aux chocs économiques. Je tiens enfin à évoquer la question des inégalités, qui tient une place très importante dans votre rapport et à laquelle nous sommes également très attachés. Comme vous le savez sans doute, le ministère de l'économie et des finances a organisé, il y a quelques semaines, une journée d'échanges et de débats Le rapport souligne, à raison, un fort creusement des inégalités depuis trente ans. Il me semble utile de rappeler que ce constat concerne essentiellement les pays anglo-saxons. La France, en effet, montre une forte résilience à ce phénomène elle se situe dans une situation plus favorable que la moyenne des pays de l'OCDE et les inégalités de revenus y sont restées stables depuis trente ans. Aussi encourageant que soit ce constat, la lutte contre les inégalités et la pauvreté n'en demeure pas moins un objectif central de la politique du Gouvernement, qui se traduit par l'adoption de plusieurs mesures phares dans la loi de finances pour 2018

Ces mesures de soutien au pouvoir d'achat, mises en oeuvre par le Gouvernement, concourent à réduire les inégalités. Le niveau de vie des ménages situés dans les trois premiers déciles de niveau de vie augmentera significativement plus que la moyenne à l'horizon 2022. À l'inverse, le niveau de vie des deux derniers déciles augmentera moins que la moyenne. Je vous invite, sur ces sujets, à vous référer au « livret du pouvoir d'achat » et au « rapport économique, social et financier », qui illustrent l'incidence des mesures décidées par le Gouvernement sur la réduction des inégalités. Mes chers

Une drôle d'impression se dégage de la lecture de son rapport, celle d'un décalage total entre l'analyse qui est faite et la réalité. La crise de 2008 était d'abord financière, avant de devenir économique. Elle est le résultat de l'éclatement d'une bulle spéculative, comme nous en avons connu d'autres dans l'histoire. Oui, les fondamentaux liés à la spéculation qui ont conduit à la crise demeurent les mêmes : il y aura évidemment d'autres crises financières dans le futur et nous nous adapterons ! Le rapport explique aussi que, paradoxalement, nous ne devrions pas craindre un nouveau krach financier, mais plutôt un embrasement social et politique, qui serait le contrecoup de la crise de 2008. Il y a là une sorte de « saut quantique », que l'on ne peut comprendre qu'en exhumant le soubassement idéologique du rapport, qui est fondé sur une grille de lecture marxiste de l'économie la finance relève de la superstructure ; l'infrastructure, ce sont les rapports de force économiques réels, qui sont entérinés par le système politique. Si la crise semble ne pas finir pour certains et que notre croissance n'est pas à la hauteur de nos principaux concurrents, c'est parce que les énergies productives demeurent bridées par toujours plus de carcans réglementaires et normatifs. La finance n'est ni un bien ni un mal, c'est une nécessité pour irriguer l'économie. À toutes les phases de son développement, une entreprise a besoin d'investisseurs. Or, depuis dix ans, les Français se sont détournés des marchés en actions, ce qui fait défaut à nos entreprises.

satisfaisant, puisque le taux d'obtention des crédits se situe à un très haut niveau historique. En revanche, sur le front des fonds propres, nous considérons qu'il existe des marges d'amélioration, en en particulier pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. C'est

répondant vingt et une fois en deux minutes ! Franchement, quel est le sens d'un tel dispositif ? Est-ce que quelqu'un pense qu'on peut sérieusement

228. « La sécurisation du système bancaire passe prioritairement et en urgence par la séparation réelle des banques de dépôt et des banques d'affaires »

des activités de nos banques entre leurs activités commerciales et leurs activités pour compte propre. Tel est le choix fait par la France.

des fonds propres des banques, comme vous le savez, nous avons déjà eu quatre séries de renforcement des régimes de Bâle, et nous arrivons progressivement dans une zone où nous sommes très à l'aise et sereins sur les bilans des banques. La

si je n'en partage que les analyses et pas les conclusions, j'estime que les travaux extrêmement complets de notre brillant collègue Collombat illustrent ce que l'on peut attendre de la délégation à la prospective obliger les responsables à anticiper l'avenir, adopter une vision prospective. Personne n'avait anticipé la crise de 2008, ni les économistes, ni les politiques. Plus grave encore, certains économistes affirmaient que le marché allait s'autoréguler et encourageaient le politique à ne pas intervenir. Or, si la crise financière, devenue économique et sociale, a pu être maîtrisée, c'est bien grâce à l'intervention du politique au niveau européen. Je partage l'analyse inquiétante selon laquelle, après dix ans de crise, la probabilité technique de réédition d'un krach du système financier d'ampleur équivalente à celui de 2007-2008 n'a pas diminué, bien au contraire. Je partage également son analyse lorsque notre collègue affirme que les responsables politiques doivent réaliser l'ampleur du danger et adopter des mesures efficaces. En revanche, il me semble dangereux d'affirmer que s'affranchir de la zone euro est la solution. Fuir plutôt que réformer et adapter ? La sortie de la crise peut également se faire non pas par plus ou moins d'Europe, mais par la construction d'une Europe différente qui prenne en compte ce risque. Le caractère systémique de la crise de 2008 est en partie dû au temps de réaction des marchés financiers, des banques et agences de notation américaines, à la limite de la fraude. Il s'agit donc d'adopter des mesures à l'échelon européen ou international permettant de donner l'alerte. En 2008, c'est bien l'Europe et une volonté politique française qui ont été la solution. Aussi, je souhaiterais savoir quelles sont les mesures d'anticipation d'une nouvelle crise que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre au niveau européen et, pourquoi pas, international. La parole est à Mme la

dans le renforcement de la régulation du secteur financier au niveau international. Il s'agit d'un enjeu international et européen. Pour des questions d'efficacité, c'est à ce niveau en effet que notre action se déploie et c'est là que nous obtiendrons des résultats. Au cours des dernières années, depuis la crise, nous avons été extrêmement proactifs pour porter des mesures ambitieuses, au sein tant du G20 que de l'Union européenne, sur le renforcement des exigences en fonds propres des banques et des assurances, sur le durcissement des règles d'utilisation des instruments financiers, y compris les produits dérivés et la titrisation, sur l'encadrement du. Nous restons Nous restons très vigilants pour que ces mesures et ces politiques avancent sur le plan international et qu'elles soient bien transposées en droit français. Nous resterons également vigilants pour que ces règles ne soient pas détricotées par certains États au plan international. Nous allons enfin travailler sur de nouveaux chantiers, en particulier au sein de l'Union européenne et au sein de la zone euro, pour promouvoir l'union bancaire. La parole

Prendre en compte la réalité est toujours pertinent, encore faut-il avoir le courage de la regarder en face. C'est ce que fait ma famille politique depuis longtemps, et, pour avoir eu raison trop tôt dans l'analyse et la dénonciation des graves dérives de l'ultralibéralisme, elle a subi et continue de subir injustement les foudres des tenants de l'idéologie mondialiste aux commandes de toutes les institutions décisionnaires. Comme le précise le rapport de M. Collombat, le terme de « populiste », que je revendique, prend la forme chez les bien-pensants de la classe politique et médiatique d'une véritable flétrissure. Les qualificatifs aussi rocambolesques qu'infamants dont nous sommes affublés servent à justifier l'exclusion du Front national du débat démocratique, quitte à manipuler, tripatouiller les modes scrutin, quitte à créer les conditions d'une crise démocratique : 13 % des voix obtenues aux élections législatives pour 1,21 % des sièges ... Les extrémistes et les ennemis de la démocratie ne sont pas ceux que l'on croit L'élection de Donald Trump aux États-Unis, le succès du Brexitet les très bons résultats électoraux des partis de droite nationale partout en Europe sont la démonstration que les peuples rejettent de plus en plus massivement le modèle, votre modèle de financiarisation de l'économie, destructeur des souverainetés et des identités. L'action du Président Macron s'apparente à un jusqu'au-boutisme qui confirme que la classe dirigeante reste sourde aux aspirations de nos compatriotes, lesquels sont chaque jour plus nombreux à réclamer plus de France. L'ancien banquier, aujourd'hui locataire de l'Élysée, impose toujours plus de déréglementation européiste, faisant la part belle aux appétits des financiers. Le fossé qui sépare la réalité des peuples et l'idéologie imposée par les extrémistes mondialistes ne cesse de se creuser. L'emblème, le moteur de ce système dont nous ne voulons plus, et qui est source de crise non seulement économique, mais aussi sociale, sécuritaire et identitaire, reste ce Moloch européiste qui dévore ses enfants européens. Comme le disait Philippe Séguin, « rien n'est plus dangereux qu'une nation trop longtemps frustrée de la souveraineté par laquelle s'exprime sa liberté, c'est-à-dire son droit imprescriptible à choisir son destin. Si charbonnier est maître chez soi, les nations, la nôtre en particulier, doivent retrouver la liberté de choisir leur destin. Nous devons travailler à établir une nouvelle confiance entre les peuples et une autre Europe, une Europe européenne, une Europe où les nations sont libres et souveraines pour mieux coopérer entre elles au service des peuples, et non plus d'un marché anonyme et déraciné. Veuillez conclure !

je me contenterai d'une réaction. Vous considérez que l'élection de M. Donald Trump et le vote en faveur du Brexit étaient un seul et même signal de rejet du monde financier et du rôle de la finance. Je vous laisse cette appréciation, que je ne comprends pas.

du pays, des entreprises et de l'ensemble de nos concitoyens, pour assurer la prospérité de tous. Le rôle du Gouvernement en matière financière est d'assurer une réglementation solide, juste, qui protège nos concitoyens. La

il existe en économie une théorie des cycles, qui peut effectivement faire craindre que, selon la judicieuse expression de Pierre-Yves Collombat, « l'histoire bégaie ». Après la longue crise, ou plutôt la succession de crises qui ont miné l'économie mondiale depuis 2007, entrons actuellement dans une phase d'embellie. Nous le savons, la croissance de l'Union européenne devrait atteindre 2,3 % en 2018. Depuis l'année dernière, tous les indicateurs économiques mondiaux passent au vert. Pour autant, la vigilance doit continuer de s'imposer, en particulier s'agissant de la possible formation de bulles ou de l'utilisation abusive de certains outils financiers. Depuis 2007-2008, les banques centrales ont mis en oeuvre des politiques exceptionnelles qui se sont traduites par des taux d'intérêt exceptionnellement bas et une liquidité surabondante. Or, selon le prix Nobel Jean Tirole- un Toulousain -, une bulle peut émerger quand le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance. Par ailleurs, quand il y a trop de liquidités, les financiers sont en quête d'actifs rentables. Le FMI s'en est inquiété à l'automne, à propos d'actifs non traditionnels comme le fameux bitcoin, qui est souvent évoqué, mais il n'est pas le seul. Je voulais évoquer également les LBO, ces rachats d'entreprises par endettement, dont les entreprises françaises sont très friandes. Je sais que le Haut Conseil de stabilité financière ainsi que la BCE ont alerté sur la hausse des emprunts bancaires et des financements par LBO, qui pourraient faire peser des risques sur la stabilité financière. La hausse des taux d'intérêt pourrait en effet fragiliser les sociétés trop endettées. Madame la secrétaire d'État, quel est votre sentiment sur ces LBO, et quelles actions préventives pourraient être envisagées

Nous exerçons une vigilance approfondie, par l'intermédiaire du Haut Conseil de stabilité financière et des pouvoirs macroprudentiels dont il dispose, sur la stabilité des marchés financiers et la valorisation des prix des actifs.

maîtrisé. La parole est à M. François Bonhomme, pour le groupe Les Républicains. Madame la secrétaire d'État, un peu plus de dix ans après le début de la crise financière mondiale, qui s'est transformée en une crise économique planétaire, toutes les leçons ont-elles été tirées, en particulier par les banques ?

Entre 2007 et 2015, elles ont doublé leur capitalisation rapportée à leurs actifs financiers. En parallèle, ces banques ont dû revoir leurs modèles pour se concentrer sur des activités compatibles avec la nouvelle donne réglementaire. Les grandes banques américaines ont mené, les premières, de lourdes restructurations qui leur ont permis de renforcer leur domination mondiale. Elles sont désormais plus grandes qu'en 2007, certes toujours un peu moins rentables, mais nettement plus que les banques européennes. Ces dernières avancent encore en ordre dispersé. La vague de publications des résultats trimestriels a confirmé que l'écart se creusait entre celles qui doivent encore achever leur restructuration, qui n'en finissent pas de payer la facture des litiges passés, et celles qui ont taillé dans le vif. L'Europe compte encore beaucoup de banques convalescentes, au bilan fragilisé par des créances douteuses. C'est notamment le cas en Italie. Dès lors, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous assurer que les produits toxiques ont été éradiqués ? Plus généralement, comment comptez-vous garantir, dans le cadre du mécanisme européen de supervision unique désormais en place,

Monsieur le sénateur, vous soulignez à raison qu'il existe des situations relativement variées au sein de la zone euro s'agissant des résultats des banques, de la situation de leur bilan,

et gérer les créances douteuses qui pourraient rester à leur bilan. J'ai mentionné voilà quelques instants une initiative et un plan d'action au niveau européen, que nous continuons à pousser afin que ces situations de créances douteuses soient peu à peu apurées. Je vous confirme que la France participe et que les autorités de la zone euro prennent toute leur part à ce travail de nettoyage qui se poursuit.

sans pour autant partager à 100 % ses conclusions. Je tiens aussi à saluer le travail de la délégation à la prospective, que je viens de rejoindre, et dont je vois tout l'intérêt et l'utilité. Madame la secrétaire d'État, j'aimerais rebondir sur un aspect évoqué dans la quatrième partie du rapport, à savoir le niveau d'investissement public dans un cadre réglementaire contraint.

la coordination et la gouvernance de l'UEM de 2012, encadrant fortement les finances publiques. Je crois d'ailleurs que les Français se réjouissent que la période où tel ou tel gouvernement laissait filer les déficits soit terminée.

nous le savons, l'investissement public a l'effet multiplicateur le plus élevé parmi les mesures budgétaires, et de nombreuses études ont montré la complémentarité qui existe avec l'investissement privé. Dit autrement, les effets sur la croissance de long terme de l'investissement public ne sont plus à démontrer. Ma question est simple, madame la secrétaire d'État : comment pouvons-nous concilier les contraintes de finances publiques, utiles et nécessaires, par ailleurs, et le financement de l'investissement public ? J'ajoute une sous-question : comment pouvons-nous, nous, parlementaires, avoir la garantie que l'investissement public soit bien fléché, donc qu'il ait un bénéfice socioéconomique non discutable ? La parole est à Mme la

de l'utilisation de ces crédits d'investissement. Il est ainsi prévu des actions pour sanctuariser les dépenses qui contribuent le plus au développement économique durable de notre pays. La parole

en octobre 2008 : « Je pense que la crise est derrière nous et que notre système économique a bien tenu. » À l'heure où moins de 2 %, 1,6 % pour être précis, des transactions financières dans le monde ont un lien avec l'économie réelle, c'est-à-dire la production de biens, de marchandises et de services pour l'humanité, nous aurions tiré toutes les leçons de la crise de 2008. La finance serait maîtrisée, régulée, contrôlée, assainie, sécurisée. Mme Couppey-Soubeyran, universitaire qui fut auditionnée par la délégation à la prospective, a dit : l'économie a souffert de la crise, le secteur bancaire pas du tout. valeur des actifs des banques françaises est passée de 7 000 milliards d'euros en 2007 à 8 500 milliards d'euros en 2014, et sans doute plus aujourd'hui. Les activités de produits dérivés dans le monde

Bien sûr, il y a eu la loi bancaire de 2013, mais tout le monde s'en est moqué. Ainsi, M. Oudéa, P-DG de la deuxième banque française, a dit devant des députés médusés, lors de son audition par la commission des finances : « Votre loi va encadrer 1 % de mon activité bancaire. » L'argent va donc beaucoup et surtout à la spéculation,

Monsieur le sénateur, vous évoquez des risques nouveaux qui s'amplifieraient depuis la crise de 2008. En effet, il y a en permanence de la créativité dans le secteur financier, comme dans tous les secteurs, mais soyez assuré que nous observons cette créativité. Nous en parlons aussi au plan international

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le rapport de Pierre-Yves Collombat fait dans le cadre de notre délégation à la prospective est un travail important. Je le remercie de nous permettre d'en débattre aujourd'hui. Dix ans après, la crise de 2008 est-elle vraiment terminée ? Selon le rapport, pas du tout ; j'apporterais pour ma part une réponse plus nuancée. La crise de 2008 n'est pas terminée, mais la situation économique s'est un peu améliorée en France. Depuis 2014, la croissance du PIB est remontée pour se stabiliser aujourd'hui autour de 1 %. Certes, c'est faible, mais c'est un début de redémarrage. Beaucoup plus inquiétant est le constat que les fondamentaux du système financier n'ont pas été réformés depuis 2008. La législation européenne n'a pas évolué. La loi bancaire de François Hollande, dont la finance était pourtant l'ennemie, n'impacterait que 0,75 % des revenus des grandes banques. Dans ces conditions, une nouvelle crise est inéluctable. Le système financier mondial actuel est naturellement générateur de bulles spéculatives. Tous les experts le disent : il y aura de nouveaux krachs. La seule chose que l'on ignore, c'est quand et de quel type d'actifs cela viendra. Pourtant, les mesures d'assainissement du système sont connues séparer les activités spéculatives et celles de financement de l'économie ; interdire les activités trop spéculatives.

dans la même entité. En revanche, dans la situation actuelle, ce sont les activités pour compte propre des banques, considérées comme spéculatives, qui sont isolées du reste du bilan des banques.

La crise de 2008 a révélé l'incapacité de la pensée économique à analyser les dysfonctionnements de la sphère financière et, par conséquent, à recommander les politiques préventives et curatives nécessaires. Aujourd'hui, les voix de Paul Romer, actuellement économiste en chef de la Banque mondiale, ou encore d'Olivier Blanchard,

l'euphorie liée aux performances économiques des années d'avant la crise aurait été moindre. Des outils de mesure intégrant des évaluations de soutenabilité- endettement privé croissant, par exemple -nous auraient donné une vision plus prudente de ces performances.

le rapport de 2017, qui devait paraître en octobre dernier, n'est toujours pas disponible. Pouvez-vous nous dire, madame la secrétaire d'État, si vous le publierez comme il se doit ? Pierre-Yves Collombat indique dans son rapport que 12 % des britanniques sont logés dans des paradis fiscaux et pratiquent des effets de levier supérieurs à 50.

Monsieur le sénateur, vous exprimez votre intérêt pour certains indicateurs qui permettraient de mesurer la richesse nationale avec une vision plus large du bien-être et de la richesse

Ce constat met en lumière l'écart grandissant entre les approches macroéconomiques et microéconomiques. En effet, cet endettement et les liquidités qu'il engendre ne semblent pas, en tout cas dans notre pays, submerger le tissu des PME. Ces dernières rencontrent toujours des difficultés pour financer leur fonctionnement et leur développement. Les règles prudentielles mises en place au niveau européen paraissent même accentuer de manière discriminatoire leurs difficultés d'accès au crédit et l'appréhension même du risque.

il est vrai qu'aujourd'hui, en France, l'accès à l'endettement, en particulier pour les PME, est plutôt bon. C'est donc plutôt du côté du capital qu'il y aurait des choses à améliorer. C'est dans ce sens que nous allons avec le PACTE.

Les Républicains. Je souhaite saluer le travail considérable réalisé par notre collègue Pierre-Yves Collombat. J'adhère pleinement à l'alerte qu'il lance quant au risque d'explosion d'un système financier virtuel. rapport le constate très justement : « Après dix ans de crise, la probabilité de réédition d'un krach du système financier d'ampleur équivalente n'a pas diminué. La plus grande crise financière de ce début de XXI siècle a en réalité commencé le 9 août 2007 en France. Ce jour-là, BNP Paribas gelait les retraits de ses clients dans trois de ses fonds d'investissement. Elle admettait ne plus pouvoir valoriser les actifs détenus dans ces fonds, car ils n'étaient plus échangeables sur les marchés. Cela démontre que cette crise était prévisible. On sait d'ailleurs qu'aux États-Unis certains experts avaient, dès 2005, anticipé la crise des et spéculé sur l'effondrement des marchés financiers. aussi que cette crise n'a atteint l'ampleur mondiale qu'on lui connaît qu'en raison de l'irresponsabilité de certaines banques et agences de notation, mais aussi à cause d'une prise de conscience internationale tardive. Il y a néanmoins toujours des signaux indicateurs de crise. Depuis cinq ans, le monde n'a connu aucune crise financière majeure, et la France va beaucoup mieux. Toutefois, les perspectives économiques de l'OFCE, dévoilées en octobre dernier, confirment ce que la presse décrit depuis plus de six mois, à savoir les potentielles causes d'une nouvelle crise : boom immobilier en Chine et en Suède, bitcoin, crise de la dette publique. La politique menée par les banques centrales a conduit les taux d'intérêt au plus bas, ce qui permet à la France de s'endetter à bas coût sans en sentir immédiatement les conséquences budgétaires. La France empruntera en 2018 un montant record sur les marchés : 195 milliards d'euros ! Inévitablement, les taux d'intérêt vont finir par remonter. Le 29 décembre dernier, Standard & Poor's envisageait un scénario catastrophe au cas où la France n'entreprendrait pas des réformes radicales. La dette atteindrait, en 2050, 166,4 % du PIB, contre 97,6 % aujourd'hui. En juillet dernier, le gouverneur de la Banque de France avait déjà donné l'alerte et insisté sur la nécessité d'une réforme des services publics. Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, nous préciser aujourd'hui si des mesures d'anticipation et de protection face à une remontée des taux d'intérêt sont prises par le Gouvernement ? La parole

vous l'avez relevé, dans le cadre de leur réponse à la crise, les banques centrales sont massivement intervenues pour permettre de financer l'économie et donc de limiter l'impact de ces crises sur la situation des populations. Elles ont abaissé leurs taux directeurs en territoire légèrement négatif afin de soutenir l'économie. Ensuite, parce que cette expansion monétaire n'a pu être suffisante, elles ont mis en oeuvre une nouvelle stratégie non conventionnelle, à savoir l'assouplissement quantitatif. Ces achats d'actifs ont permis d'influencer plus directement les taux de long terme, qui guident les décisions d'investissement. Dans le contexte actuel, les grandes banques centrales devront trouver le bon équilibre pour soutenir la reprise économique et éviter les excès financiers. Même si la reprise économique se poursuit, l'inflation reste faible, ce qui amènera probablement les banques centrales à ne durcir que très graduellement leur politique. Toutefois, elles seront également attentives aux prises de risque croissantes des acteurs financiers et pourraient chercher, conjointement avec les autorités prudentielles, à éviter des excès qui pourraient être source de crises futures. S'agissant de la façon dont nous anticipons leurs changements de politique ou l'évolution graduelle de leur politique, ce point a bien été pris en compte dans la trajectoire des finances publiques. Vous pourrez noter que le Gouvernement a d'ores et déjà anticipé une augmentation graduelle des taux d'intérêt et son impact sur nos charges financières. La M. Didier Rambaud, pour le groupe La République En Marche. Madame la secrétaire d'État, les analyses d'économistes le montrent et la presse spécialisée s'en fait l'écho régulièrement : la réglementation et la supervision du secteur bancaire n'épousent pas totalement les contours des différents canaux du financement de l'économie.

les, qui n'affecte pas l'ensemble de ces fonds. Je voudrais aussi rappeler que, selon le Conseil de stabilité financière, les sommes gérées par le représentaient en 2015, à l'échelle mondiale, environ 92 000 milliards de dollars, soit l'équivalent de la moitié du système bancaire traditionnel.

vous l'avez noté, depuis la crise, le système bancaire parallèle joue un rôle croissant dans le financement de l'économie réelle, en particulier en apportant de nouveaux outils de financement aux entreprises. Compte

le Conseil de stabilité financière s'en sont saisis. La France joue un rôle moteur pour pousser ces discussions dans les instances internationales nous participons aux groupes de travail sur ce sujet et nous proposons des mesures concrètes pour permettre de mieux comprendre et de mieux réguler ces activités.

c'est tout de même à partir d'un segment étroit- les crédits immobiliers aux particuliers -que s'est propagée une véritable thrombose des marchés financiers, mal qui a touché, par ricochet, l'ensemble des secteurs financiers. Il nous faut détricoter le problème, dans notre diversité. On sait quelles mesures durent être prises pour redonner un peu de liquidité à des activités bancaires frappées par la méfiance réciproque et la chute libre des cours de bourse. Ces derniers mois, malgré la politique bienveillante de la BCE en termes de création monétaire, la France connaît une situation paradoxale. Les

Concernant les ménages, la croissance de l'endettement atteint près de 6 % en glissement annuel, avec une augmentation marquée des crédits à la consommation et des crédits liés à l'habitat. De notre point de vue, cet endettement des ménages, s'il a permis de de porter une partie de l'activité économique en 2017, est aussi porteur de risques pour la solidité du secteur financier dans les années à venir. En effet, les taux d'intérêt réels associés aux emprunts sont sans commune mesure avec la progression du pouvoir d'achat.

Monsieur le sénateur, je ne reviendrai pas sur mon constat initial : nous ne rejoignons pas vos vues sur le rôle de la finance dans l'économie.

2008, justement, l'année même où la finance mondiale entrait dans une crise d'une ampleur exceptionnelle, naissait une technologie qui semble capable, à terme, de transformer le monde de la finance et de l'argent. Je veux parler du bitcoin. Le bitcoin est ce que l'on appelle une crypto-monnaie : une monnaie numérique qui a pour particularité de ne pas être soumise au contrôle des États ou d'un quelconque tiers. L'Histoire avance. Hier, l'or, les billets ; aujourd'hui, les chèques, les cartes bleues ; demain, le bitcoin ? On voit que nos paiements quotidiens sont de plus en plus dématérialisés. Ce n'est peut-être qu'un début. Le bitcoin, en effet, va beaucoup plus loin en n'existant que sur le réseau informatique et en se passant d'intermédiaire. Certains y voient une bulle ; d'autres, une révolution comparable à l'imprimerie, à la micro-informatique ou à l'Internet. Le passionnant rapport de la délégation sénatoriale à la prospective sur les perspectives de la finance mondiale n'intègre ni l'émergence du bitcoin et des autres crypto-monnaies ni leur influence potentielle sur le système financier mondial. En outre, ces nouvelles monnaies peuvent également révolutionner le rapport entre politique et finance. Nous devons le prendre en compte et l'anticiper. En complément à ce passionnant rapport, le Gouvernement peut-il nous apporter son point de vue et son éclairage sur le phénomène du bitcoin et des crypto-monnaies, phénomène qui va peut-être changer l'Histoire ? La

Cela dit, aujourd'hui, la capitalisation totale de ces actifs, qu'on appelle, pour la plupart, des « crypto-monnaies », représente environ 700 milliards de dollars.

de même pour l'information et les risques qui se manifestent pour les investisseurs non professionnels

Je retiendrai une de ses conclusions, celle qui m'apparaît comme la plus préoccupante : « la probabilité d'un nouveau crash du système financier comparable à 2007-2008 ». La question n'est donc plus de savoir si ce crash aura lieu, mais quand il aura lieu. Ainsi, les fonds publics déversés au moment de la crise n'auront pas suffi à faire prendre conscience des indispensables mesures à prendre pour nous prémunir des errances et des inconséquences du monde de la finance. Le constat fou que seulement 10 % des échanges boursiers sont en rapport avec l'économie réelle est la démonstration que ce système, sans contrôle, sans régulation imposée, peut nous mener au désastre. La technocratie financière a pris le pouvoir depuis trop longtemps c'est au pouvoir politique de lui reprendre. Pour cela, profitons de ce qui a commencé à faire ses preuves, certes avec des imperfections : je veux parler des conférences mondiales sur l'environnement, les COP. Il est indispensable que les pays qui se sont retrouvés pour échanger, proposer et décider dans les COP environnementales fassent de même sur les questions financières et fiscales. C'était une proposition d'Éric Bocquet et d'autres ; je m'y rallie volontiers. En effet, nous n'imaginons pas que la France ait les capacités d'agir seule, tant il est vrai que la finance n'a pas de frontières. Nous ne pouvons pas, pour paraphraser le général de Gaulle, faire notre petite soupe, à petit feu, dans notre petit coin ! Portons cette initiative de COP financière et fiscale internationale Sinon, c'est l'égoïsme habituel qui risque de prévaloir et de nous conduire, une fois encore, à une errance financière majeure et à la catastrophe économique et sociale qui, malheureusement, risquerait d'en découler.

On ne peut pas exclure de nouvelles crises. Ce qui est sûr, c'est que, progressivement, nous avons appris des événements qui ont eu lieu et nous avons mis en place des systèmes

que c'est bien à un niveau international et européen que doivent se prendre les bonnes décisions. La parole est à M. Michel Raison, pour le groupe Les Républicains.

Bel exemple que le financement du crédit immobilier « à la française », dont la remise en cause serait très préjudiciable. Il repose sur trois spécificités : des taux majoritairement fixes, une analyse sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur et une garantie reposant souvent sur le cautionnement plutôt que sur l'hypothèque. Si ce modèle français avait prévalu aux États-Unis en 2007, la crise des et les terribles images des emprunteurs expropriés n'auraient certainement pas existé. Soyons un peu chauvins ! Les épargnants et les emprunteurs français sont plutôt bien protégés aujourd'hui. Ces caractéristiques doivent donc être préservées. Or les travaux internationaux menés par le Comité de Bâle pourraient remettre en cause le crédit immobilier « à la française Le Sénat, dans sa grande sagesse, a adopté à l'unanimité en 2016 une résolution de notre excellent collègue Didier Guillaume visant à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle. Nous lancions alors une alerte sur les risques que pourraient engendrer ces nouvelles règles. Depuis, l'accord de Bâle a été signé et il doit être transcrit en droit européen. Madame la secrétaire d'État, ma question portera donc sur l'avenir de cet accord, dont une partie des recommandations a mené l'économie mondiale presque dans l'impasse. J'espère fermement que vous ne laisserez pas ces règles s'imposer à nous et que vous affirmerez, comme le Sénat a su le faire en 2016, que la régulation financière doit s'imposer pour protéger les Français. Le courage politique, ce n'est pas que des décisions imposées aux Français en politique intérieure ; c'est aussi à l'extérieur !

est traité le système français de crédit immobilier dans le cadre prudentiel international de Bâle qui va être transposé en droit européen.

de la pratique des banques françaises soit bien prise en compte. Nous sommes relativement confiants ; en tout cas, cette exigence est bien comprise au plan européen. Nous avons donc intégré ce sujet. C'est

cela a été dit -le fonctionnement du capitalisme financier transnational et les difficultés systémiques passées et, hélas, certainement à venir. Je voudrais revenir sur le financement de l'économie réelle par les banques. Je devrais plutôt parler de non-financement, tant la part consacrée à ce financement est faible par rapport à l'ensemble des transactions financières réalisées par les opérateurs financiers. Le rapport pose bien la question : « À quoi sert réellement le marché financier ?

la poursuite de pratiques risquées. Risquées pour qui ? Pour nos États et pour nos populations, car aujourd'hui, au vu des mesures qui sont prises, nous sommes toujours, en cas de crise grave, dans une situation où les risques pris seront couverts par la puissance publique. Quelle est donc l'utilité de ce marché financier Le rapport cite, à titre d'exemple, la somme de 32 000 milliards de dollars d'échanges de titres à Wall Street sur un an, alors que le besoin annuel de financement des entreprises n'est que de 250 milliards de dollars par an, soit moins de 1

et d'orientation de l'épargne vers les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Toutes les dispositions prévues ne sont pas encore prises. Une première série

menée, après deux ans, me semble-t-il, en tout cas dans le courant du quinquennat, une évaluation de l'impact de ces mesures gouvernementales sur l'économie réelle. La

L'histoire peut-elle bégayer indéfiniment ? Je ne le crois pas. Le politique peut-il, dans ce cas, jouer le rôle de l'orthophoniste ? Je le crois profondément. En 2007-2008, notre monde a connu la pire crise financière de son histoire depuis celle de 1929. Malgré tout, un certain nombre d'acteurs du système financier continuent à considérer que le marché est le seul et unique instrument de régulation. Personnellement, je crois dans le libéralisme économique, dans la possibilité pour chacun de réussir, pour chaque entreprise de se développer sans entrave ; je crois dans un marché libre et créateur de richesses. Mais je ne crois pas à l'effacement du monde politique face à l'économie. Je ne crois pas que notre rôle soit de ramasser les débris après une crise ni que nous soyons élus pour nous ranger aux prédictions et aux recommandations d'un système imbriqué auquel on ne peut pas toujours faire confiance. Notre rôle n'est-il pas au contraire d'imaginer l'économie de demain, une économie respectueuse de l'environnement, consciente de l'enjeu social, libre mais régulée, une économie, surtout, au service de l'économie réelle J'ai été consternée, à la lecture de ce rapport, par un chiffre : 5 % seulement de l'activité bancaire servent au financement des entreprises ; 5 %, mes chers collègues ! Qu'avons-nous tous collectivement raté pour constater de tels chiffres aujourd'hui ? Le laisser-aller en matière économique a engendré une défiance profonde à l'égard des États, des entreprises, de l'économie, à l'égard d'un système qui donne le sentiment de se liguer contre les intérêts des citoyens. Les discours populistes prospèrent sur l'incapacité des décideurs publics à faire changer les choses. Promenez-vous, mes chers collègues, dans les rues de chacune de nos villes. Vous entendrez sûrement l'un de nos concitoyens vous dire que, en votre qualité d'élu, vous n'avez aucun pouvoir en matière économique. Et peut-on le blâmer pour cela ? Je ne le crois pas. C'est collectivement l'image que nous renvoyons depuis des décennies : une classe politique atone face au monstre spéculatif, impuissante face à la destruction de l'économie de notre pays, résignée face à l'étiolement de son pouvoir.

Elles sont cruciales : on n'avancera que si l'Allemagne et la France unissent leurs forces dans le même sens. est le souhait exprimé par le Président de la République, annonçant, main dans la main avec la Chancelière allemande, une position commune de nos deux pays sur le sujet crucial de la zone euro d'ici à mars prochain.

Sur ces points concrets, nous voulons enregistrer des progrès à très court terme, en 2018. Au-delà, la France oeuvrera pour défendre une transformation en profondeur et ambitieuse de la zone euro, en particulier par la mise en place d'une capacité budgétaire

Il est défendu par le ministère du travail, mais l'ensemble du Gouvernement est extrêmement mobilisé. Nous parlons de formation professionnelle, d'apprentissage, de réforme des lycées professionnels, également, avec Jean-Michel Blanquer. L'accès à une main-d'oeuvre qualifiée, à un encadrement de qualité, partout sur le territoire et surtout pour tous les métiers, est extrêmement important. Certains métiers sont aujourd'hui en tension

en 1637 éclatait le premier krach boursier, celui des tulipes, aux Pays-Bas. Au plus fort de la bulle spéculative, le prix d'un bulbe de tulipe équivalait à quinze fois le salaire annuel d'un artisan. Et puis, brutalement, les cours se sont effondrés. Cette histoire de la spéculation, nous la connaissons : elle s'est répétée, comme l'a rappelé mon collègue Collombat dans son rapport d'information, à travers de nombreuses crises financières mondiales. Elle se répète encore aujourd'hui, avec une fréquence d'ailleurs accentuée ces dernières années.

La poussée fulgurante de cette monnaie virtuelle, créée à l'issue de la crise des en 2009, a connu des records en décembre. Objet de toutes les spéculations et de tous les fantasmes, mais aussi phénomène de mode, le bitcoin a vu son cours augmenter de 1 000 % en un an, atteignant les 11 500 dollars l'unité, avant de violemment rechuter. Quelle volatilité ! La non-traçabilité des opérations, sa valorisation irrationnelle, sa nature même, qui est dématérialisée, font du bitcoin une valeur insaisissable, et donc dangereuse dangereuse pour les épargnants qui achètent cet actif, dangereuse parce qu'il peut facilement être utilisé pour financer des activités illicites- fraude fiscale, blanchiment, terrorisme, trafics en tous genres. Le bitcoin nous donne des sueurs froides, non pas tant parce qu'il menace directement l'équilibre du système financier mondial, mais parce qu'il échappe au contrôle des États, des banques centrales et des institutions financières. La spéculation sur le bitcoin est symptomatique des dérives du fonctionnement de notre économie. La mise en place d'un cadre réglementaire efficace relatif au bitcoin, et plus largement aux crypto-monnaies, ne pourra se faire que une vaste coopération internationale. À raison, M. le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, prend ce sujet au sérieux et a souhaité que le G20 s'en saisisse lors de son prochain sommet. Pas plus tard qu'hier, il a confié à l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France, Jean-Pierre Landau, une mission sur les crypto-monnaies. Ma question est donc la suivante : quelles sont les différentes pistes de réflexion avancées pour faire évoluer la réglementation et ainsi protéger nos concitoyens face au bitcoin ? La parole

position complètement fermée par principe. Tel est l'équilibre sur lequel nous avons proposé à Jean-Pierre Landau de travailler. Mes

L'ordre du jour appelle le débat sur la prise en charge des mineurs isolés, organisé à la demande du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. citoyen et écologiste. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'orateur du groupe

Ses pupilles jonglent dans tous les sens. Tout dans l'environnement de notre bureau semble lui susciter une crainte. [ ...] Il a beaucoup de mal à décrire sa vie dans son pays. À chaque fois, le voyage jusqu'en Europe arrive en trombe dans son esprit. [ ...] « Tout se mélange : les rebelles sur la route au Nord-Mali la traversée du désert du Sahara, dans un pick-up surchargé ; les travaux d'esclaves dans le bâtiment, dans chaque ville-étape, pour trouver l'argent nécessaire à la poursuite de la route [ ...]. Moussa se souvient des sept mois à Gourougou. Tous les migrants la connaissent, cette [ ...] forêt, juchée sur la montagne qui surplombe l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. [ ...] Sept mois à vivre dans des tentes de fortune, à se faire déloger par les policiers marocains, à tenter de survivre. Et surtout, sept mois à attendre le bon moment pour [ ...] tenter d'escalader la triple barrière de six mètres de haut pour mettre un pied sur le sol européen. [ ...] « Moussa a échoué six fois, avant de réussir. [ ...] six fois les barbelés qui mordent, six fois les matraques, six fois le refoulement à la frontière algérienne. Six fois l'espoir qui explose au sol en tombant. Au moment où il le raconte, il touche machinalement le haut de sa main gauche, marquée d'une cicatrice. La barrière a sorti les griffes et mangé la chair. Sur le haut de son crâne aussi.

ce qu'a écrit Rozenn Le Berre, alors éducatrice auprès des mineurs isolés étrangers, dans son livre, témoignage de 547 jours passés avec les mineurs isolés étrangers. Je vous invite à prendre connaissance des dizaines d'autres récits poignants de ces vies en sursis, de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes qu'on évalue et pour lesquels on décide : mineur ou majeur, protégé ou expulsé, un toit ou la rue, la vie ou l'exil. Avant de traiter du sujet sous l'angle des chiffres et de la loi, il est aujourd'hui plus que nécessaire de se confronter à ces réalités, à ces histoires personnelles qui font notre histoire commune. La vague de cynisme qui surplombe le sommet de l'État ces dernières semaines n'en est pas digne. Non, il n'est pas question de « bons sentiments », mais il est question de sentiments tout court, et pour ainsi dire d'humanité, de solidarité, de fraternité. il est nécessaire de repenser aux causes à l'origine de ces migrations : aujourd'hui les guerres, les crises économiques dans lesquelles notre responsabilité n'est pas exempte ; demain les sinistres liés au réchauffement climatique et la nouvelle vague de réfugiés qu'il faudra bien prendre en compte. Pour l'heure, et pour en venir aux chiffres, que se passe-t-il réellement ? Sur le million de personnes très vulnérables identifiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, seules 200 000 ont été prises en charge. La France est le quinzième pays d'accueil des réfugiés, derrière de nombreux pays qui sont loin d'avoir notre puissance économique. Ces chiffres nous amènent à relativiser la réalité de la situation l'Europe est loin d'être la première destination des réfugiés, les migrations s'établissant davantage entre pays du Sud et, au sein de l'Europe, la France est loin de prendre sa part. notre pays ne joue pas pleinement son rôle pour protéger et accueillir les réfugiés, à commencer par les plus vulnérables d'entre eux : les enfants. Dans ce cadre, la politique migratoire envisagée par M. Macron et le Gouvernement apparaît plus qu'inquiétante ; en témoignent les circulaires Collomb du 20 novembre et du 12 décembre derniers visant à organiser un tri entre migrants migrants et dans les centres d'hébergement d'urgence. Ces circulaires, vous le savez, ont suscité un tollé dans le monde associatif, mais pas seulement, comme l'illustrent les nombreuses voix qui se sont exprimées ces derniers jours ; et nous sommes solidaires du recours contre la circulaire Collomb porté devant le Conseil d'État par une vingtaine d'associations de défense des étrangers et de lutte contre l'exclusion. Cette approche de la politique migratoire de notre pays, qui porte atteinte aux droits humains, est plus que préoccupante, et dans ce cadre nous pensons aux plus vulnérables qui viennent nous demander refuge, aux mineurs isolés- nous les appellerons ainsi et non pas « mineurs non accompagnés », termes repris de l'usage des institutions européennes par nos politiques pour, semble-t-il, édulcorer le sens des mots, cette expression étant bien plus proche de la réalité. Contrairement à ce que laissent entendre certains cris d'orfraie poussés à droite, il n'existe pas de statut juridique propre aux mineurs isolés étrangers. Ces derniers se trouvent donc à un croisement, relevant à la fois du droit des étrangers et, au titre de l'enfance en danger, du dispositif français de protection de l'enfance qui ne pose aucune condition de nationalité. C'est le statut d'enfant qui devrait prévaloir, conformément aux engagements de la France au titre de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pourtant, à l'issue du dernier congrès des départements de France, Édouard Philippe a annoncé qu'il entendait, entre autres, transférer la prérogative d'accueil des mineurs isolés étrangers à l'État, remettre en cause la présomption de minorité et la présomption d'authenticité des actes lors de l'orientation des mineurs vers l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Si les départements sont à juste titre préoccupés,

que les mineurs isolés étrangers ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des mineurs et jeunes majeurs accueillis dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, soit environ 18 000 sur 325 000. Ceux que reçoivent notamment les associations telles que Médecins du Monde renvoient incontestablement à des profils d'enfants souvent très abimés, physiquement ou psychiquement. Rappelons également que la mise à l'abri n'est pas systématique. Lorsqu'elle a lieu, elle se fait dans des conditions très contestables, parfois dans des hôtels insalubres, sans accompagnement ni suivi par un éducateur. Enfin, le premier accueil est uniquement dédié à l'évaluation de l'âge et à l'isolement de jeunes qui ne sont pas en mesure d'être évalués. Voilà pour le cadre

il est nécessaire de mettre fin immédiatement à l'enfermement, sous quelque forme que ce soit, de tous les mineurs étrangers, aux frontières comme sur le reste du territoire, et au contraire mettre en oeuvre une mise à l'abri inconditionnelle pour les personnes se déclarant mineurs isolés étrangers, comme le prévoit la loi au nom du respect de la présomption de minorité. Ensuite, il est urgent de mettre fin aux tests osseux, et plus globalement aux ingérences du ministère de l'intérieur dans le dispositif d'évaluation médicale, et de restaurer la tutelle du ministère chargé de la santé. Sur ce point, rappelons, comme s'accorde à le dire l'ensemble de la communauté scientifique, qu'il n'existe aucune méthode objective et fiable pour évaluer la minorité d'une personne. En cas de persistance d'un doute, celui-ci doit profiter au jeune. Tout examen médico-légal doit être interdit. La santé qui soigne n'a pas vocation à être un outil à expulsion. Enfin, à l'opposé des solutions envisagées par le Premier ministre, nous pensons, comme le suggèrent plusieurs syndicats, dont le Syndicat de la magistrature, qu'il est temps d'instaurer un dispositif de prise en charge des mineurs isolés étrangers juridiquement contraignant pour les conseils départementaux et de sanctionner les départements récalcitrants, notamment pour que le nombre de places d'hébergement en foyer éducatif et en famille d'accueil soit augmenté, accompagné des postes de travailleurs sociaux afférents, le tout sans discrimination en matière de financement entre enfants français et étrangers. Il est primordial de revenir au droit commun de la protection de l'enfance impliquant l'abrogation du dispositif dérogatoire de la loi du 14 mars 2016 pour prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien entendu, ce retour au droit commun devrait s'accompagner d'un financement important de l'État pour abonder les budgets gérés par les départements et du développement d'outils opérationnels de soutien aux professionnels chargés des mineurs étrangers isolés. Dans cette logique, il semblerait cohérent national de financement de la protection de l'enfance créé par la loi du 5 mars 2007. Enfin, comme le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, nous mettons en garde le Gouvernement « sur les risques que pourrait comporter une telle réforme, notamment au regard des engagements internationaux de la France, au premier rang desquels la Convention internationale des droits de l'enfant. » Ratifiée par la France en 1990, celle-ci s'applique à tous les enfants, sans considération de nationalité ni d'origine ethnique ou sociale.

En conclusion, la prise en charge des mineurs isolés étrangers en France est insuffisante, et ne répond pas à leurs besoins fondamentaux et à la protection qui leur est due. Or les propositions faites ces derniers mois, que ce soit par le biais du rapport d'information sénatorial publié en juin dernier ou par l'Assemblée des départements de France, soutenue par le Premier ministre, ne feront qu'aggraver la situation. Il est notamment absolument nécessaire d'abandonner l'idée d'un dispositif dérogatoire au droit commun qui tendrait à considérer ces jeunes mineurs isolés d'abord comme des étrangers avant d'être des enfants à protéger. C'est là un angle primordial du débat ; j'espère qu'il guidera vos questions, mes chers collègues, et vos réponses, madame la garde des sceaux.

pour traduire la réalité de cette question des mineurs isolés, comme vous avez choisi de les appeler, madame la sénatrice, mais pour lesquels je reprendrai la terminologie plus habituelle de « mineurs non accompagnés Le contexte, de ce point de vue, a changé en quelques années. En 2013, le nombre de personnes qui se présentaient comme mineurs non accompagnés ne dépassait pas quelques milliers.

un dispositif, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, de répartition des mineurs non accompagnés entre les différents départements de notre pays. C'est également une loi, une loi, je tiens à le réaffirmer au regard de vos propos, madame la sénatrice, qui vise à garantir à ces mineurs isolés, ou non accompagnés, les mêmes droits qu'à tout autre enfant présent sur le territoire. C'est bien le statut d'enfant qui prime toute autre considération en l'espèce, la difficulté tenant évidemment à la manière de déterminer la minorité de l'enfant. quelques chiffres, dans un premier temps, expliquant en partie les tensions que nous connaissons sur ce dispositif et qui sont ressenties sur l'ensemble du territoire. L'augmentation du nombre d'arrivées a été extrêmement importante jusqu'à la fin de l'année dernière, avec une hausse très rapide à partir du mois de juin 2017. Ce fait a engendré de réelles difficultés pour répondre au besoin de mise à l'abri durant l'été ; il a également été à l'origine d'attentes plus longues pour la mise en oeuvre du dispositif d'évaluation, ou encore pour les prises en charge effectuées à l'issue du dispositif d'orientation. Du 1 janvier au 31 décembre 2017, le nombre de mineurs confiés aux départements par décision judiciaire s'est élevé à 14 908, soit 85 % d'augmentation par rapport à l'année 2016.

Par ailleurs, 13 000 mineurs non accompagnés étaient pris en charge dans les services de l'aide sociale à l'enfance au 31 décembre 2016. À titre de comparaison, ils étaient 10 000 l'année précédente. Je veux également insister sur un autre point : les chiffres que je viens de vous communiquer ne reflètent pas la réalité des mises à l'abri, du premier accueil en urgence des personnes qui se déclarent mineurs non accompagnés. En croisant les données des derniers rapports, notamment de Mme la sénatrice Doineau et de M. le sénateur Godefroy, de Mme la députée Bagarry, ainsi que les données de l'Agence de services et de paiement gérée par le ministère des solidarités et de la santé, le nombre de personnes se déclarant mineurs non accompagnés et devant être mis à l'abri, puis évalués par les départements a atteint, cette année, 25 000. Les

J'en viens au dispositif légal, dont je vous rappelle très simplement comment il fonctionne. Dès qu'un mineur non accompagné arrive sur notre territoire, il est mis à l'abri

département ait une charge équitable ou, en tout cas, des obligations équitables par rapport à ces mineurs. Malgré les difficultés que cela pose, je pense que nous pouvons nous féliciter de ce système. Le code civil impose aux magistrats du parquet et aux juges des enfants de saisir la cellule nationale gérée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui va formuler une proposition d'orientation vers un autre département ou

Le procureur de la République ou le juge des enfants prendra ensuite sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Cette clé de répartition est calculée en fonction des données démographiques et tient compte

Quelles sont les difficultés rencontrées sur l'ensemble de ce dispositif ?

Les difficultés tournent autour des points suivants, que j'énumère devant vous brièvement : la très forte augmentation du nombre de personnes qui se déclarent mineures ; la saturation totale

l'absence d'harmonisation des pratiques en matière d'évaluations de la minorité réalisées sur le territoire national-

Face à ces difficultés réelles, les enjeux sont cruciaux. Il s'agit de fiabiliser et d'harmoniser les procédures d'évaluation,

il nous faut porter remède. Le Président de la République s'est engagé, lors du conseil des ministres du 12 juillet dernier, à ce que la situation des mineurs non accompagnés soit de nouveau envisagée dans sa globalité. À la suite de cela, le Premier ministre a signé a signé avec Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, une lettre de mission destinée aux corps d'inspection de l'administration de la justice et des affaires sanitaires et sociales pour que soit engagée une réflexion,

base des éléments qui nous seront proposés, sur lesquels je reviendrai dans quelques instants, nous devrons de nouveau établir un plan de prise en charge des mineurs non accompagnés. Je vous remercie, monsieur le président,

ce lundi, dans un communiqué de presse, l'Assemblée des départements de France exprimait, une nouvelle fois, son inquiétude quant à l'absence de réponse de l'État sur la prise en charge des mineurs non accompagnés, et ce malgré les engagements du Premier ministre du mois d'octobre dernier. En effet, l'État s'était engagé à prendre en charge l'évaluation et l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineures entrant dans le dispositif jusqu'à ce que la minorité soit confirmée. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités et opte pour une attitude humaniste à l'égard des migrants mineurs qui traversent les mers, bien souvent à leur corps défendant. En vertu de l'article 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces enfants exilés ont « droit à une protection et une aide spéciales de l'État. » Le phénomène des mineurs qui deviennent majeurs au cours de la procédure d'évaluation entache profondément notre rôle d'assistance. des solidarités et de la santé souhaite promouvoir une « logique d'investissement social » dans le cadre d'un plan de lutte contre la pauvreté des jeunes, il me paraît nécessaire d'élargir cette idée cette idée à la question des mineurs isolés, dont le sort ne peut être abandonné aux seules collectivités locales ou aux associations. Dans la Sarthe, par exemple, leur prise en charge est en constante augmentation. Le département consacre près de 4 millions d'euros à la prise en charge des 171 mineurs recensés, et l'on assiste à la saturation des structures d'accueil disponibles, comme partout en France. Au-delà de la question financière, primordiale, à l'appui de l'excellent rapport de mes collègues Élisabeth Doineau et Jean-Pierre Godefroy, je souhaite aborder la problématique spécifique, mais essentielle, de la formation de ces mineurs après seize ans. De sérieux dysfonctionnements ont été constatés quant à la délivrance d'autorisations provisoires de travail nécessaires au suivi de formations professionnelles généralement dispensées par un Ainsi, ma question porte sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour réaffirmer le droit inconditionnel des mineurs non accompagnés à obtenir une autorisation provisoire de travail et pour faciliter l'accès de ces jeunes à la formation professionnelle, qui est une

notamment pour les enfants qui ne pouvaient accéder à des formations professionnalisantes du fait d'un défaut de documents d'identité. Elle a clarifié les autorisations provisoires dont ceux-ci peuvent avoir besoin

substituer au département, ainsi que la région, qui en a la compétence. Il faudrait, quatrièmement, simplifier l'obtention des titres de séjour pour les mineurs réfugiés, afin que ceux-ci puissent travailler dès leur majorité lorsqu'ils sont diplômés. Je vous remercie, madame la garde des sceaux, de l'intérêt que vous voudrez bien porter à l'examen de nos propositions.

nous le savons, la politique, c'est d'abord un combat sémantique. Et ce combat prend ici toute son ampleur lorsque le politiquement correct évoque des MNA, des mineurs non accompagnés, alors que la réalité voudrait qu'on les nomme des EMC, des étrangers mineurs clandestins. Entre 2010 et la fin de 2016, leur nombre est passé de 4 000 à 13 000, pour dépasser les 25 000 à la fin de 2017 et atteindre, cela a été dit, 40 000 en 2018. Sans compter que ces chiffres restent largement sous-évalués puisqu'ils ne comptabilisent pas les jeunes dont les démarches sont en cours. Le véritable scandale réside dans le fait que 70 % de ces jeunes clandestins sont en réalité majeurs. Prouvez-le ! Les entretiens censés déterminer si une personne est mineure relèvent de la fumisterie. Or les mineurs, non soumis aux règles de séjour des étrangers, ne sont pas expulsables. Dont acte. Une simple déclaration de leur part les rend éligibles à l'aide sociale à l'enfance conseils départementaux qui en assument la charge ; une charge qui aura représenté un milliard d'euros en 2016, 2 milliards en 2017. La prise en charge annuelle d'un mineur isolé étranger représente 60 000 euros par an. Pour le département des Bouches-du-Rhône, le coût est de 20 millions d'euros pour les contribuables. Les clandestins peuvent, eux aussi, dire : « Merci Martine présidents de droite de conseil départemental, ce coût doit être supporté non plus par les départements, mais par l'État. Autrement dit, plutôt que de faire payer le contribuable, on fera payer ... le contribuable. Voilà une belle idée, comme dirait Laurent Wauquiez. Et c'est le Conseil de l'Europe qui nous met le coup de grâce, je le cite : « Les jeunes migrants ne doivent pas être soumis contre leur gré à des examens médicaux visant à déterminer leur âge, et doivent, en cas de doute, être considérés comme des mineurs. » Eh oui ! Cette présomption d'innocence constitue, de toute évidence, un nouvel appel d'air à l'immigration clandestine. Nous devons rétablir les frontières, démanteler les filières de passeurs, utiliser tous les moyens adéquats pour savoir si ces clandestins sont mineurs ou pas, et enfin expulser les clandestins adultes. Le problème est identifié et les mesures efficaces existent. La seule question, madame la ministre, est de savoir si vous aurez le courage de les appliquer.

Le quart de ces migrants sont des Soudanais et des ressortissants d'Afrique francophone : Ivoiriens, Maliens, Guinéens. Un nombre important d'entre eux

Aucune expulsion n'est possible une fois que l'enfant mineur est entré sur notre territoire. L'accueil est inconditionnel dans le cadre de la protection de l'enfance, sans considération de l'origine ni de la nationalité. Il est prévu un encadrement strict du recours aux tests osseux, assorti d'une présomption de minorité. Nous soutenons l'élaboration d'un référentiel pour harmoniser les pratiques d'évaluation de l'âge en garantissant à la fois un regard bienveillant et pluridisciplinaire. Nous sommes donc à la fois très stricts et très vigilants sur les obligations légales et sur la coopération

madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l'accueil des étrangers en France fera prochainement l'objet de débats approfondis. Au sein de cette vaste question, les solutions à apporter aux limites du système actuel d'accueil des mineurs non accompagnés pourraient en particulier, me semble-t-il, faire l'objet d'un consensus minimal. Au-delà des critiques externes qui se multiplient aujourd'hui, au sein de la Cour européenne des droits de l'homme, du Comité des droits de l'enfant de l'ONU ou de la part d'associations comme l'UNICEF, la situation sur notre sol d'errance administrative de ces jeunes, parfois encore des enfants, est contraire à plusieurs principes de notre droit l'irresponsabilité des mineurs, leur droit à la scolarisation, à un hébergement et à l'accès aux soins. En octobre dernier, le Premier ministre a déclaré que « l'État assumera l'évaluation et l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineurs entrants [ ...] jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée Doineau et notre ancien collègue Jean-Pierre Godefroy soulignent que le dispositif de l'ASE n'est pas dimensionné pour répondre à ces demandes de nouvelle nature et de nouvelle ampleur. Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes demandant à bénéficier de l'ASE a été multiplié par 2,5. Les cinq jours d'hébergement d'urgence remboursés pour l'évaluation de la minorité représentent une durée bien inférieure aux délais réels observés dans différents départements. Malgré la bonne volonté des conseils départementaux, certains jeunes se trouvent sans solution d'hébergement dans ce laps de temps, ce qui les expose à un risque d'exploitation par des réseaux de traite. ce stade, les pistes envisagées par le Gouvernement ? Ne serait-il pas possible de mettre en place des plateformes interterritoriales, financées par l'État, rassemblant des personnels dûment formés à ces problématiques particulières, permettant une meilleure prise en charge de ces personnes le temps de l'évaluation de minorité et avant

entre les départements et éviter que les ordonnances de placement provisoires pour poursuite d'évaluation quant à la minorité ou l'isolement ne soient prises en charge que par les départements, en attendant que la minorité ou la majorité soit déterminée.

Il est difficile pour ces collectivités locales de faire face à une présence accrue de mineurs isolés. Dans mon département, les Bouches-du-Rhône, 577 sont recensés, chiffre qui a plus que doublé. de l'ASE ne sont pas égaux face à la situation en fonction de leurs difficultés propres et du nombre de mineurs isolés à prendre en charge, qui varie d'un département à l'autre, et ce malgré les mécanismes de péréquation.

Aussi, madame la ministre, je souhaite savoir où en est la réflexion entre l'État et les départements pour une meilleure articulation, voire une meilleure répartition de la prise en charge de ces mineurs isolés. En effet, M. le Premier ministre avait donné quelques assurances à ce sujet lors de son déplacement à Marseille pour le congrès de l'Assemblée des départements de France. Ne pourrions-nous pas maintenir l'expertise des départements en la matière, dans leur rôle de protection de l'enfance, et convenir simplement d'une participation financière de l'État

l'État rembourse au département l'équivalent de cinq jours à 250 euros, soit 1 250 euros. Selon l'Assemblée des départements de France, la dépense pour 2016 et pour l'ensemble des départements se serait élevée à 155 millions d'euros,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 21 décembre dernier, je me suis rendue au centre pour mineurs non accompagnés ouvert par Médecins sans frontières à Pantin. J'y ai passé la matinée à dialoguer avec l'équipe de professionnels qui les accueille, les informe et les oriente, et à observer ces jeunes hommes épuisés par l'exil et la vie dans la rue depuis leur arrivée sur notre territoire. La sérénité qui règne là est frappante, mais laisse peu à peu place à la révolte. Révolte de constater la faillite totale de l'État dans son devoir de protection de l'enfance. Révolte à l'écoute des récits de ces jeunes et face à la maltraitance des institutions à leur égard. Un garçon de quatorze ans s'est présenté ce matin-là au centre. Il dormait dans la rue depuis plusieurs jours. Il s'était soumis au dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers pour être pris en charge. Or, dès le guichet, il lui avait été notifié qu'il n'était pas mineur et ne pouvait entrer dans aucun dispositif, ce, à l'évidence, en violation de notre droit et de nos engagements internationaux. En octobre dernier, lors d'un déplacement dans la vallée de la Roya, j'ai assisté, à la gare de Menton-Garavan, à une tentative de renvoi en Italie d'une jeune fille de seize ans. Les forces de l'ordre, supposées la protéger, l'escortaient pour s'assurer qu'elle reprenne le train. ma question est simple : que compte faire le Gouvernement pour que soient enfin respectés, sur notre territoire, les lois françaises, le droit international et le plus élémentaire des devoirs, celui de protéger tous les mineurs ? Madame la sénatrice, votre question est à la fois juridiquement pertinente et humainement très sensible. Elle est liée à la minorité ou à la majorité de la personne qui se présente sur notre territoire. C'est bien dans cette reconnaissance de minorité ou dans cette déclaration de majorité

C'est le rôle de l'État d'accueillir dignement une personne étrangère sur notre territoire, de lui assurer la protection correspondant à son statut, de s'assurer que les titres qu'elle présente sont authentiques, de déterminer enfin son âge. Il nous faut donc mettre en place des dispositifs d'accueil et un processus de prise en charge spécifique adapter les dispositions législatives ; clarifier la question des coûts. » De ces mots du Premier ministre ressort à la fois l'exigence éthique que nous devons avoir, et à laquelle nous avons souscrit

Face à cette situation, le Premier ministre a annoncé que l'État assumerait, à la place des départements, l'évaluation et l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineures, et ce jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée. Cependant, et comme plusieurs orateurs avant moi l'ont rappelé, une grosse partie du financement revient toujours aux conseils départementaux, la protection de l'enfance. En effet, comme vous le savez, la prise en charge peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Ainsi, plusieurs problèmes se posent, notamment la saturation des structures d'accueil, l'impossibilité d'anticiper la progression des dépenses budgétaires, ou encore l'urgence de situations particulières et complexes. L'accueil de ces jeunes non accompagnés n'est pas remis en question, mais certains départements semblent plus concernés que d'autres. Et c'est précisément parce que ces jeunes doivent être pris en charge dans de bonnes conditions que les départements demandent plus de garanties à l'État, pour des personnes qui se présentent de plus en plus sans document d'identité, ce qui complexifie l'évaluation de la minorité. Dans leur rapport de juin 2017, les sénateurs Élisabeth Doineau et Jean-Pierre Godefroy soulignaient déjà la nécessité de revoir le processus d'évaluation. Si les agents de l'aide sociale à l'enfance, chargés de l'accueil et de l'accompagnement des mineurs isolés, font de plus en plus preuve de compétences spécifiques- linguistiques, géopolitiques ou sociologiques le juge des enfants semble rarement tenir compte de ces évaluations initiales, qui sont systématiquement remises en cause lorsqu'un jeune déclaré majeur engage un recours les associations. Au-delà de l'aspect financier, c'est bien une amélioration du dispositif que les départements sont en droit d'attendre. Ne pensez-vous pas qu'une formation partagée, cohérente et adaptée de l'ensemble des acteurs permettrait des décisions mieux comprises et un accueil plus serein des mineurs isolés ? La parole est à Mme la garde des

La parole est à Mme Laure Darcos, pour le groupe Les Républicains. Madame la garde des sceaux, je suis consciente d'être redondante par rapport aux précédentes interventions de certains de mes collègues, mais cela montre la gravité de la situation de part et d'autre. Notre pays accueille chaque année toujours plus de mineurs étrangers privés de la protection de leur famille. C'est une réalité qu'il faut appréhender avec objectivité, sans esprit partisan ni volonté polémique. Oui, nous devons protection à ces mineurs, comme nous y engage la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont la France est signataire. Oui, nous devons mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour faciliter leur parcours migratoire et leur insertion future, et les aider à devenir des citoyens éclairés et responsables. En revanche, nous devons lutter avec une extrême fermeté contre les filières migratoires faisant venir sur notre territoire des adolescents ou des jeunes adultes à des fins strictement économiques, voire d'exploitation s'apparentant à une traite des êtres humains. Dans mon département, l'Essonne, la situation devient particulièrement préoccupante, avec l'arrivée non régulée et difficilement maîtrisée d'un très grand nombre de mineurs non accompagnés, plus de 600 en 2017. Les établissements dédiés à la protection de l'enfance sont débordés, les travailleurs sociaux, formés avant tout pour apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique à l'enfance en danger, sont contraints de mettre en oeuvre des actions d'accompagnement social et éducatif qui ne relèvent pas de leur compétence première. Le conseil départemental assume néanmoins toutes ses responsabilités, y compris financières- plus de 30 millions d'euros de dépenses budgétaires en 2017 -et vient en appui des associations, qui font un travail de terrain tout à fait remarquable. L'actuelle organisation fait cependant courir aux départements et à leurs présidents des risques juridiques majeurs, notamment de nature pénale. Ces derniers ne disposent pas, en particulier, du pouvoir de réquisitionner les logements nécessaires à la mise à l'abri des mineurs concernés, contrairement à l'État, qui se refuse certaines fois J'en appelle donc au bon sens pour traiter ce problème critique et souhaite, madame la ministre, des mesures fortes de la part de l'État, qui doit agir sans tarder pour mieux contrôler les évaluations et permettre aux départements de recentrer leur action sur les jeunes les plus vulnérables. La parole

Marche. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans notre pays, cela a été dit, on dénombre plus de 25 000 mineurs isolés étrangers, concentrés principalement à Paris, dans le Nord-Pas-de-Calais et la Seine-Saint-Denis. S'il est devenu habituel d'occulter la question ultramarine, je me suis donné comme mission de la rappeler systématiquement au bon souvenir de notre assemblée et des différents gouvernements qui se succèdent. À Mayotte et en Guyane, la problématique des mineurs étrangers isolés dépasse largement la politique d'aide sociale à l'enfance relevant des conseils départementaux, par ailleurs fragiles financièrement. Le contexte géographique de ces deux départements les soumet à une pression migratoire intense, qui intéresse les ministères de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères, et qui rend irréalisable une quelconque péréquation.

Aussi, madame la garde des sceaux, je souhaite tout d'abord savoir quand les départements d'outre-mer, notamment la Guyane et Mayotte, pourront au minimum se voir appliquer les dernières dispositions législatives, particulièrement le dispositif national de mise à l'abri et, mieux encore, pour compenser l'absence de péréquation, bénéficier bénéficier d'un prolongement de la prise en charge financière au-delà des cinq jours. Ensuite, est-ce que le Gouvernement envisage de mettre en place une solution pérenne en engageant une véritable coopération avec les pays avoisinants et en développant une réflexion interministérielle sur ce sujet ? Marche. Monsieur le président, madame la ministre,

M. Dominique Watrin, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Madame la ministre, j'étais lundi à Calais avec les principales associations d'aide aux migrants pour faire le point sur la question des mineurs isolés qui échouent dans cette ville dans l'espoir d'un passage clandestin au Royaume-Uni. Selon ces associations, ces mineurs représentent entre 40 % et 60 % des 700 migrants actuellement présents dans le Calaisis, soit entre 300 et 400 jeunes. La plupart seraient admissibles au droit d'asile ou au rapprochement familial s'ils avaient accès au sol britannique. Mais le déplacement de la frontière anglaise de Douvres à Calais du fait des accords du Touquet les en empêche. Lors de la fermeture de la jungle de Calais, plus de 700 dont nombre de mineurs isolés, avaient été admises en Grande-Bretagne, et cela en 24 heures, alors que beaucoup d'entre eux étaient préalablement bloqués à Calais depuis des semaines, vivant dans la lande une expérience souvent traumatisante. Je veux aussi adresser un démenti à tous ceux qui instrumentalisent ces situations pour en pour en rendre responsables les associations, lesquelles apportent pourtant aide et réconfort à ces mineurs et sauvent heureusement l'honneur de notre pays. Madame la ministre, le président Emmanuel Macron va rencontrer demain Mme Theresa May. Quels moyens va-t-il enclencher pour obtenir l'admission en urgence des mineurs isolés qui vivent dangereusement à Calais ? Je vous rappelle que quatre d'entre eux ont perdu la vie en un mois sur la rocade. Je pense aussi à ces jeunes qui sont dans les griffes des réseaux de passeurs, victimes parfois des pires trafics d'êtres humains. Quelles mesures pour obtenir l'examen rapide des dossiers des autres demandeurs d'asile et pour gérer, de façon efficace et humaine, sur le long terme, le passage légal vers la Grande-Bretagne, dans le respect des accords internationaux dont nos deux pays sont signataires ? Le renforcement des mesures sécuritaires a montré ses limites ; on peut rajouter des kilomètres de grillage, cela ne changera pas beaucoup la situation. Il faut renégocier les accords du Touquet, en remettant la frontière là où elle était. Plus généralement, c'est un autre partenariat qu'il faut

Je souhaite vous interpeller sur trois points et vous faire deux propositions pour ce qui concerne Mayotte. Tout d'abord, l'amélioration de l'attribution des délégations d'autorité parentale aux proches peut faciliter le tutorat par les familles des enfants

Enfin, quels sont les moyens financiers que l'État pourrait accorder de manière exceptionnelle au conseil départemental de Mayotte pour une mise en place rapide des prérogatives de la collectivité au titre de l'ASE,

2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale qui s'applique à Mayotte, ainsi qu'aux régions Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté ? Deuxièmement, comment pourrait-on faciliter la conclusion d'accords bilatéraux entre les Comores et Mayotte, sur le modèle signé avec la Roumanie en 2003 ? La parole

le passage à la majorité d'un jeune qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a besoin d'un accompagnement spécifique, en particulier pour le droit au séjour et l'intégration dans notre société ? La parole est à Mme la garde des sceaux.

d'enjeux organisationnels, financiers et diplomatiques, ce sont pour la plupart des enfants et des adolescents seuls dont il est question. Leur périple pour arriver en France a été douloureux, dangereux, violent. Il est des témoignages qui sont insupportables à entendre. Ce phénomène, qui s'est considérablement accéléré ces derniers temps, est dramatique et humainement insupportable. Il laisse souvent désemparés tous les acteurs institutionnels. Ce phénomène migratoire semble s'installer dans la durée ; nous ne pourrons donc plus nous contenter de réponse au coup par coup et dans l'urgence. Aujourd'hui, ils sont près de 50 000 à être attendus dans notre pays. Leur nombre a plus que doublé en deux ans. Le coût de leur prise en charge par les conseils départementaux a été l'an dernier de plus de 1 milliard d'euros. Dans le département des Ardennes, leur nombre a été multiplié par trois au cours de l'année passée. Si les départements ont des compétences et des responsabilités bien précises en matière d'aide sociale à l'enfance, il n'en va pas de même pour les mineurs non accompagnés, dont la mise à l'abri et la prise en charge relèvent de la politique migratoire de l'État. Toutefois, dans l'urgence, les départements ont dû se substituer à l'État. Or, aujourd'hui, ceux-ci n'ont plus les moyens en personnel, en locaux et tout simplement financiers pour faire face. Concernant ces mineurs, l'État a désormais pris conscience de la situation, et il y a un souhait de la part de tous les acteurs institutionnels de bien faire. Il importe donc désormais qu'une répartition équitable de la charge financière entre l'État et les départements devienne réalité. Il faut aussi mettre en place une gestion partagée par l'État et les départements d'un dispositif permettant d'assurer un accompagnement adapté aux situations spécifiques des requérants. cette dramatique question des mineurs migrants- osons le mot ! -doit être abordée avec la plus grande fermeté à l'égard des passeurs, odieux raquetteurs sans scrupules, et avec la plus grande dignité et humanité envers ces jeunes enfants et adolescents. madame la garde des sceaux, mes chers collègues, c'est bien une politique migratoire d'ensemble qu'il faut construire en France et coordonner au niveau de l'Union européenne.

Dans mon département, la Haute-Loire, le nombre de ces jeunes mineurs est évalué à 110, dont 86 ont été pris en charge en 2017. Le dispositif actuel de l'aide sociale à l'enfance, qui place ces jeunes sous la responsabilité du président du conseil départemental, permet de répondre à leurs besoins vitaux, mais ne favorise pas toujours un accompagnement social à visée d'intégration et d'insertion professionnelle. En effet, ces jeunes mineurs sont malheureusement souvent accueillis dans des structures hôtelières, à défaut d'autres solutions plus adaptées. À travers mon expérience professionnelle de directeur d'établissement accueillant ces jeunes mineurs isolés, j'ai pu constater à la fois la motivation et le souhait de ces derniers d'être rapidement autonome grâce à un parcours de formation assez court ou en alternance de type apprentissage. Ces jeunes sont en général très mobilisés, et le récit de leur parcours en témoigne. Ils disposent, pour un certain nombre d'entre eux, de réelles capacités d'adaptation dans des métiers tels que l'industrie, le bâtiment ou l'hôtellerie, secteurs d'activité qui aujourd'hui rencontrent de véritables difficultés de recrutement. De très bons résultats sont aujourd'hui constatés à travers certaines expériences apportant une réponse plus adaptée, notamment à partir de la transposition du dispositif HOPE- hébergement, orientation, parcours vers l'emploi -mis en oeuvre par l'AFPA. Il s'agit en effet de travailler prioritairement sur la qualification et les compétences de ces jeunes sur certains types d'emploi. Madame la garde des sceaux, certes le dispositif ASE permet de répondre partiellement à l'accueil de ces mineurs non accompagnés, mais n'est-il pas urgent de réfléchir, dans le cadre d'une véritable politique migratoire, et compte tenu du fait que ces flux ne vont qu'augmenter à l'avenir, à la mise en oeuvre généralisée d'un dispositif spécifique plus adapté à la prise en charge des mineurs non accompagnés ? Cela permettrait à la fois à l'État de procéder à la phase d'évaluation- cela a déjà été évoqué -et aux départements, en lien avec les partenaires locaux de leur choix, de développer un accompagnement principalement axé sur l'insertion et la formation professionnelle.

antérieur. L'éducation nationale a le devoir, pour ces enfants comme pour tous les autres, à la fois de leur enseigner les fondamentaux du système éducatif, comme le français, et de les insérer le plus rapidement possible dans une scolarité classique.

non accompagnés qui ont été recensés en 2016, un nombre qui ne cesse de croître et qui devrait être largement dépassé en 2017. Ces mineurs sont très fragilisés physiquement et psychologiquement après une errance souvent longue et douloureuse. Les inquiétudes sur les conditions dans lesquelles nous les accueillons sont multiples. L'évaluation de leur situation et de leur minorité est trop brutale sans qu'ils aient été préalablement mis à l'abri pour un temps de répit. Elle est incertaine, comme cela a été souligné précédemment. Le nombre de solutions adaptées reste faible ; ils sont trop nombreux à l'hôtel où ils demeurent pour l'essentiel livrés à eux-mêmes, la plupart d'entre eux n'ont même pas accès aux soins. Une fois accueillis, beaucoup sont privés de scolarisation. Ainsi, en Seine-Maritime, sur un groupe de 80 mineurs suivis, seule une quarantaine étaient scolarisés, 25 restaient en attente de place et une quinzaine étaient laissés sans solution. Il n'y a aujourd'hui qu'un seul agent au rectorat pour répondre à leur situation, et rien n'est prévu pour ceux qui sont illettrés et les non-francophones. Le Premier ministre a annoncé que l'État assumerait désormais l'évaluation et l'hébergement d'urgence de ces mineurs. Certes, ce geste peut être perçu comme bienvenu pour aider des départements saturés. Toutefois, il appelle à la vigilance, car il serait dangereux que l'accueil des mineurs non accompagnés soit organisé dans le cadre des politiques migratoires. Ces jeunes doivent être considérés comme des enfants et non comme des étrangers ; ils ne peuvent être accueillis dans les mêmes dispositifs que les adultes et doivent bénéficier de notre système de protection de l'enfance sans discrimination.

Le discours peut être volontariste, mais la situation actuelle n'est pas digne des valeurs de la France. Pouvez-vous nous indiquer quels moyens le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour assurer une réponse humaniste, apporter un soutien significatif aux départements et favoriser l'inclusion scolaire de ces jeunes ?

selon une étude de l'ADF, étaient de 40 jours en moyenne en 2017, avec des pics à 180 jours dans certains départements, alors que seules 5 journées sont remboursées aux départements. lorsque le Premier ministre propose que l'État reprenne à sa charge la période d'évaluation, c'est plus qu'un « geste », si je peux me permettre de reprendre votre expression : c'est à la fois une volonté

importante. Le Premier ministre l'a aussi clairement dit, l'État ne fait pas de l'accueil des enfants une politique migratoire. Nous parlons bien des enfants

Au total, à ce jour, plus de 250 mineurs non accompagnés sont confiés au département. Or, après une décision de majorité, nous observons aujourd'hui des jeunes qui déposent parfois un recours contre les conseils départementaux et des jeunes déclarés majeurs qui se déplacent dans différents départements afin d'essayer d'obtenir le statut de mineur. On assiste alors également à un phénomène de changement d'identité. Ce nomadisme a un coût financier important, puisqu'il mobilise les services départementaux les uns après les autres, ainsi que la police aux frontières. Sur la seule année 2017, le budget consacré par le département de la Charente-Maritime était de 5 millions d'euros. Le budget prévisionnel pour 2018 affiche 6 millions d'euros. En dépit de ces chiffres, la Charente-Maritime n'est pas dans le peloton de peloton de tête des départements les plus touchés par ce phénomène- vous les avez rappelés tout à l'heure. Vous n'ignorez pas que cette situation inquiétante intervient bien sûr dans un contexte de baisse de dotations aux collectivités territoriales. Bien sûr, la convention internationale relative aux droits de l'enfant existe, de même que les droits de l'homme et l'humanité, mais la politique migratoire de la France ne peut être la même que celle qui a été pratiquée par le passé et doit se discuter au niveau européen ; vous en avez convenu tout à l'heure. Le contexte a changé, et nous devons prendre acte de ces mutations. Sur la question des mineurs non accompagnés, il faut effectivement agir en adulte responsable. Avons-nous les moyens de l'exigence éthique exprimée par le Premier ministre et que vous venez de rappeler, madame la garde des sceaux ? En attendant, le Gouvernement entend-il mener une action dans le but de permettre la mise en place d'un fichier biométrique, afin de mettre fin aux phénomènes de fraude à l'état civil, de changements d'identité et d'assurer un véritable suivi de ces jeunes qui sont entrés dans notre pays ? La parole est

la mission d'inspection demandée par le Premier ministre réfléchit à cette question. La demande de réévaluation

troisième possibilité serait de rendre l'évaluation opposable dès lors qu'elle a été réalisée. Nous réfléchissons sur ces différents points, en nous appuyant chaque fois sur la police aux frontières pour les questions d'identité, car elles sont aussi importantes.

comme nombre d'anciens conseillers départementaux. L'enfant est une personne vulnérable qu'il faut bien sûr encadrer, soigner et protéger

Les jeunes qui demandent la prise en charge sont âgés et saturent le dispositif. S'ils sont vraiment majeurs, il faut les épauler en mettant en place d'autres dispositifs. Mais il ne faut pas faire reposer ce problème uniquement sur les épaules de l'aide sociale à l'enfance. L'augmentation exponentielle des jeunes supposés mineurs dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, comme dans tous les autres départements, entraîne une explosion des coûts d'accueil d'urgence. Le prix de l'aide sociale à l'enfance est de 166 euros par jour en France, ce qui correspond à 60 000 euros par enfant et par an. C'est un lourd problème financier qui fragilise toute la protection. Les services du département du Nord évaluent à 30 % le nombre de jeunes adultes parmi les demandes d'accueil des mineurs non accompagnés. Les juges, faute de moyens et de preuves, se rangent à la présomption de minorité et condamnent les départements à payer des astreintes pour les loger. Les départements sont donc obligés de les accueillir au sein de maisons d'enfants, afin de ne pas payer ces astreintes. Dans le même temps, des enfants sont en danger au sein de leur famille- j'insiste sur ce point. Faute de place, ils sont contraints de courir le risque de maltraitance au sein de leur famille. dans mon département du Nord, où 200 mineurs en danger ne peuvent être admis dans les centres d'accueil. Madame la garde des sceaux, ces chiffres sont aussi dramatiques que les autres

c'est non seulement pour prendre acte de la partie régalienne de ce dispositif, mais aussi pour soulager financièrement les départements et donc leur permettre réellement, dans le cadre de l'ASE,